L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

articles additionnels après l'article 2. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement

Aujourd'hui, le maire est trop souvent dans l'incapacité de faire respecter les actes relevant de ses prérogatives. En cas de non-respect d'une de ses décisions administratives, notamment en matière de police,

à affaiblir son autorité et sa légitimité. Comment le premier magistrat de la commune peut-il demeurer légitime et crédible auprès de ses administrés s'il doit attendre parfois plus d'une année pour faire appliquer ses décisions ? Cet amendement vise à doter le maire d'un moyen rapide, direct et dissuasif pour agir à l'égard des contrevenants. Il s'agit de garantir que l'ensemble de ses arrêtés soient respectés dans un délai de trois jours à compter de leur publication sous peine du déclenchement d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 500 euros.

est à Mme Toine Bourrat. En l'état actuel du droit, les maires des communes concernées par un plan d'exposition au bruit sont soumis à des contraintes spécifiques justifiées par les caractéristiques propres à leur géolocalisation. Parmi celles-ci figure la restriction des conditions d'attribution de permis de construire dans les zones jouxtant des aéroports

il n'est pas autorisé à demander aux pétitionnaires de lui fournir d'autres pièces justificatives. Cet amendement tend donc à lui attribuer tous les moyens nécessaires à l'obtention de pièces justificatives prouvant que la création de logements situés dans une zone aéroportuaire est en conformité avec les principes du code de l'urbanisme. amendement a pour objet d'augmenter le montant des amendes sanctionnant la réalisation de travaux illégaux. Un nombre important de contrevenants qui réalisent des travaux en méconnaissance des règles pourtant définies par le code de l'urbanisme sont condamnés à verser des sommes dérisoires au regard du préjudice commis.

l'astreinte dont peut être assortie la mise en demeure adressée à un contrevenant réalisant des travaux illégaux soit consignée jusqu'au jugement définitif. Il s'agit de limiter les pratiques dilatoires des contrevenants ayant un puissant effet dissuasif et assurant, en cas de recours, une effectivité minimum des actes pris par le maire. Quel

Celui-ci vise à permettre à l'autorité compétente pour délivrer des autorisations d'urbanisme de demander tout document permettant de vérifier que le projet respecte le plan d'exposition au bruit.

aux activités aéronautiques, aux activités industrielles et commerciales autorisées dans la zone ou à l'activité agricole. Toutefois, le maire est déjà en mesure de vérifier ces éléments, que ce soit à travers la qualité du demandeur ou la notice du permis de construire, sans qu'il soit nécessaire de produire des pièces supplémentaires.

bal de la CTAP. Cette instance de consultation territoriale à l'échelle régionale fait l'objet d'un intérêt certain. De nombreux amendements, extrêmement différents, voire contradictoires,

que les différentes collectivités territoriales et l'État savent se mettre autour d'une table, travailler et agir intelligemment, en complémentarité, quand la

semaines, d'éminents représentants de très grandes associations d'élus qui avaient trouvé notre idée absolument saugrenue, voire

je me permets d'intervenir ici pour tempérer l'enthousiasme que l'on prête aux Bretons sur le sujet.

à l'ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences » ? L'institutionnalisation de cette conférence territoriale de l'action publique

un lieu de dialogue et de convergence pour aller vers plus de cohérence, mais il faut laisser le soin à l'ensemble des collectivités

Mme la ministre.

à l'issue de ce dialogue informel, mais bien organisé tout de même, il y a un vote des collectivités territoriales.

aura, indépendamment de la CTAP, la capacité à agir intelligemment et collectivement pour l'intérêt général.

autocentrée, chacun tourné vers ses propres compétences, ce qui rend impossible toute construction interterritoriale. Or, pour délivrer des services publics, pour mettre en place des politiques structurantes, il est nécessaire d'avoir une réflexion interterritoriale.

nous permettons des délégations de compétences entre collectivités et des délégations de compétences « ascendantes », c'est-à-dire des EPCI vers les départements ou les régions.

l'avis du Gouvernement ?

pour la commune ou pour l'intercommunalité, mais de faire en sorte que le bloc communal fonctionne ; c'est complètement différent ! Je vais

au sein de l'intercommunalité, afin que celle-ci puisse déléguer de façon ascendante une compétence totale ou partielle. En écho à ce qui vient d'être

sont autorisées « avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale », c'est-à-dire la majorité qualifiée.

de transferts de compétences de l'intercommunalité vers d'autres échelons de collectivités territoriales, comme la région ou le département. C'est la raison pour laquelle il faut considérer la vision intercommunale, donc celle des composantes de l'intercommunalité, car c'est un transfert de compétences qui a déjà été effectué des communes vers l'intercommunalité. Si ces

avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale

l'avis de la commission

l'avis de la commission ?

Merci